auront certainement noté que la commission spéciale a ouvert la conservation des embryons au secteur privé. J'avais demandé qu'il soit précisé qu'il s'agit du secteur privé à but non lucratif, désormais appelé Espic depuis la loi HPST.

Si la mesure d'autoconservation des gamètes est défendue par le Gouvernement et partagée par un certain nombre de sénateurs, je le redis, il n'a jamais été dans ses intentions d'y associer une campagne d'incitation, en particulier à l'intention des jeunes femmes. Nous ne sommes confrontés ni à un déficit d'offre ni à un besoin d'augmenter le nombre d'établissements autorisés- je pense notamment aux établissements qui pourraient avoir pour objectif de recruter le plus de candidates possible.

Par ailleurs, nous espérons que les gamètes non utilisés seront orientés, si la personne concernée y consent, vers le circuit du don. L'exercice de l'activité de conservation dans les établissements publics ou privés à but non lucratif facilitera, par construction, le transfert des gamètes vers le secteur du don. Je suis assez confiant sur le fait que les limites posées par le projet de loi, notamment en termes de bornes d'âge- même si nous nous sommes opposés sur ce point lors des discussions de la fin de la matinée -, seront de nature à empêcher une inflation des demandes et un débordement des centres spécialisés. Nous travaillons d'ores et déjà avec les professionnels de la procréation, notamment du secteur public, pour mieux anticiper la mise en oeuvre de ces mesures. Pour l'ensemble de ces raisons, nous souhaitons revenir au texte initial du Gouvernement, ce que prévoit cet amendement.

ou tissus germinaux pour procéder à un arrêt de leur conservation. Ce délai est le même qu'il s'agisse d'une conservation sur indication médicale ou hors indication médicale. Nous proposons que ce délai de conservation avant destruction en l'absence de réponse au courrier de relance annuel soit réduit à cinq ans si la conservation des gamètes est effectuée en dehors des indications médicales. La démarche de conservation de gamètes hors indication médicale étant volontaire, aucun argument ne pourrait justifier l'absence de réponse au courrier concernant le devenir des échantillons conservés en dehors du décès de la personne.

Depuis 2004, seuls les établissements publics et privés à but non lucratif peuvent être autorisés à pratiquer cette activité ; 34 établissements de ce type l'exercent effectivement sur le territoire. Par conséquent, il n'existe pas de déficit d'offre de soins

avez voté l'ouverture aux établissements privés à but lucratif de la possibilité de procéder à l'autoconservation. Ces

modifié. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

avec la possibilité de révéler soit des informations non identifiantes, soit l'identité exacte du donneur, soit les deux.

étendu, de sorte qu'il ne connaît pas non plus le nom du donneur de gamètes, tout comme ce dernier ne connaît pas l'identité des enfants qu'il a pu engendrer par son don. Cette situation a créé un malaise chez un certain nombre d'enfants issus du don, qui s'en sont fait l'écho médiatiquement- vous les avez sans doute déjà entendus -et qui ont fait part de la nécessité pour eux, pour leur construction psychique, de connaître l'identité de la personne qui avait donné

en droit français.

L'enfant né du don sollicitera la possibilité de connaître le nom du donneur ou ses données non identifiantes et le donneur sera à son tour sollicité pour faire droit ou non à cette demande, évidemment avec un accompagnement de l'un comme de l'autre. Je précise que nous avons étendu ce dispositif

Là aussi, la question est délicate et sensible. Doit-on considérer que le principe de l'anonymat du don entre en contradiction avec le droit de l'enfant d'avoir accès à ses origines ? Nous avons entendu plusieurs associations d'enfants nés par PMA. Pour certaines d'entre elles, pouvoir disposer de ces données est indispensable indispensable à la construction individuelle. Cette impossibilité est pour l'heure source de souffrances. Pour d'autres, au contraire, cette quête d'identité, qui peut également être source de souffrances et de déception, n'est en rien utile, tant ces enfants font primer la parentalité sociale sur le biologique. ont grandi et évolué dans une famille où ils ne ressentent pas le besoin d'en savoir plus sur leur géniteur. Bien sûr, je distingue, dans les deux cas, le fait d'informer son enfant de son mode de conception du fait d'accéder à ses origines. On ne sait que trop combien les secrets, les non-dits, peuvent être lourds de conséquences dans une famille, notamment en termes d'histoire individuelle. Je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut révéler dès son plus jeune âge à l'enfant son mode de conception.

tel qu'il a été réécrit par la commission spéciale, est satisfaisant : d'un côté, au moment du don, le donneur doit exprimer son consentement à fournir ses données non identifiantes en cas de demande de l'enfant à sa majorité de l'autre, lors de la demande de l'enfant- donc, au minimum, dix-huit ans après le don -, on sollicite le donneur pour savoir s'il accepte ou non de révéler son identité. Cela revient à considérer que les données non identifiantes sont les plus importantes et que l'identité du donneur peut être davantage source de troubles pour l'équilibre de la famille. Toutefois, je m'interroge également sur le fait que, en fonction du choix

revient ainsi sur le principe d'anonymat opposable aux enfants nés d'un don de gamète ou d'embryons, principe issu de la loi du 29 juillet 1994 et conservé lors de la révision de la loi Bioéthique de 2011. Les personnes nées d'un don auront simplement la possibilité, si elles le souhaitent et à condition qu'elles sachent qu'elles sont nées d'un don, de saisir une commission dédiée, à l'instar de ce qui se passe en Suède, en Autriche, en Norvège, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Finlande ou encore en Allemagne. Les pays conservant un anonymat absolu, comme la France, se trouvent de plus en plus isolés en Europe. Pourquoi lever ce voile ? Une fois encore, la pratique n'a pas attendu la loi. Le principe d'anonymat devient obsolète en raison du développement des technologies génétiques, lesquelles permettent d'avoir facilement accès à ses données génétiques et, donc, de retrouver, éventuellement, son géniteur.

non pas dans une quête affective ou à la recherche d'une famille, mais à la recherche d'une partie de leur histoire et de leur identité. Par ailleurs, cela évite le risque de consanguinité et permet de connaître ses antécédents médicaux. C'est un changement culturel assumé

n'est pas un parent de substitution ; il est un donneur de gamètes. Il s'agit simplement de permettre à ceux qui le désirent d'avoir accès à un morceau non négligeable de leur identité, cela répond à un besoin profond chez certains enfants nés d'un don. C'est donc un droit à l'identité, qui permet que chacun puisse avoir un accès aux informations permettant d'établir quelques racines de son histoire et les circonstances de sa naissance. L'ignorance des origines est souvent une cause de souffrances mise en lumière par des psychiatres, des psychanalystes et des sociologues.

Ainsi, tous les enfants pourront avoir accès aux données non identifiantes du tiers donneur, notamment aux antécédents médicaux, mais seuls les donneurs qui le souhaitent donneront leur identité aux enfants issus de leur don.

n'est pas remis en cause. Ce principe s'exerce entre un donneur et un receveur. Or l'enfant né d'un don de gamètes constitue un tiers, tant à l'égard du donneur qu'à l'égard du receveur. l'anonymat du don n'est pas remis en cause dans le système que nous proposons. Cela dit, effectivement, les pédopsychiatres confirment la difficulté de se construire dans le secret et la frustration suscitée par ce qui s'apparente à un trou noir dans l'histoire et le récit des personnes nées de PMA avec don. le Gouvernement prévoit de compléter le cadre actuel de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, en accordant aux seules personnes conçues par don anonyme qui le souhaiteront un droit d'accès à des informations relatives au donneur, y compris à son identité. Il n'est pas question de permettre au donneur ni au receveur de connaître l'identité l'un de l'autre, ni au moment du don ni ultérieurement, et personne ne fait ni ne doit faire l'amalgame entre un père et un donneur

peu par provocation- vous m'en excuserez -, qu'il vaut mieux, dans ce cas, préserver les fameux secrets de famille ; ne bougeons pas, ne créons pas une inégalité, un supplice de plus pour ces enfants.

que les anciens donneurs ne seraient pas sollicités, mais qu'ils pourraient, sur leur initiative, se manifester auprès de la commission s'ils étaient favorables à la communication de leur identité aux personnes nées de leurs dons qui en feraient demande. Votre commission spéciale a adopté un amendement ayant pour objet de prévoir que l'on recherche les anciens donneurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir ; nous avions prévu

cela ne veut pas dire qu'il y a moins de donneurs. Je me permets de vous rappeler à cet égard que l'ouverture de la PMA aux femmes ne nécessite,, que des spermatozoïdes et non des gamètes féminins. Or il n'existe aujourd'hui aucune tension sur les dons de spermatozoïdes ; depuis que les personnes n'ayant pas eu d'enfant ont le droit de donner leurs gamètes, il n'y a plus de pénurie de spermatozoïdes. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, quelques points sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Vous le comprendrez, je serai particulièrement tenace sur la question de l'identité du donneur, parce que cela me semble fondamental pour les enfants de ce pays qui seraient nés d'un don.

D'ailleurs, les généalogistes vous le diront, ils sont très sollicités par des gens qui ont largement dépassé l'âge de l'adolescence et des crises post-pubertaires. Il est Il est assez légitime, quand on est un être humain, de se raccrocher à ses ascendants, à son histoire, à ses racines. Il y aura, pour cela, quoiqu'en dise la loi,

qui consiste à ne pas créer deux catégories différentes : les enfants qui auraient le droit de connaître leurs origines et ceux qui ne pourraient pas exercer ce droit parce que le donneur

et on va appliquer un dispositif qui me semble terriblement incompréhensible. Je n'ai pas de réponse à mes questions, mais j'aimerais bien que vous nous aidiez à résoudre toutes ces contradictions, monsieur le secrétaire d'État.

L'un des sujets qui nous préoccupe est de savoir si l'on va intégrer à ces progrès de la médecine et de la conception l'idée que la filiation peut-être multiple. Issue d'un projet parental, c'est une filiation sociologique : un couple

la fiction de la biologie dans un couple qui n'a qu'une filiation sociologique constitue une erreur. Je rejoins ce qu'a dit notre collègue Gérard Longuet : l'enfant, arrivé à sa majorité,

demander ou non l'identité de leur donneur. Mesdames, messieurs les sénateurs, une fois encore, je ne peux que vous encourager à vous mettre à la place de l'enfant au moment d'exprimer votre vote.

à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Le groupe socialiste et républicain défend le principe d'accès aux origines de l'enfant né d'un don.

origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées d'un don. L'amendement n° 292, présenté par le Gouvernement,

nous serions en porte-à-faux avec le contrat moral que nous avons passé avec eux au moment de leur don sous un régime spécifique de non-consentement pour l'accès aux origines. Pour

pour lui demander son accord, mais sans aucune garantie pour la suite. Pour notre part, nous voulons que la demande puisse recevoir une réponse. Nous avons choisi non de partir de la demande des personnes, mais d'organiser une vaste campagne d'information à l'attention du grand public pour proposer à tous ceux qui ont fait des dons dans les Cécos

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à supprimer l'obligation du recueil de consentement de l'autre membre du couple dans le cadre du nouveau droit d'accès aux origines.

Par ailleurs, il est nécessaire d'adapter le don de gamètes aux évolutions de la société et de le sécuriser en permettant au seul donneur de gamètes de révoquer son consentement. Vous avez assorti votre dispositif d'une vérification que l'autre membre du couple est toujours en couple avec le donneur au moment de la demande d'accès à l'identité de ce dernier. Rendez-vous compte de la complexité que cela peut représenter

Quel est le système le plus juste ? Quel est le système le plus égalitaire ? Quel est le système qui heurte le moins ? Aucun système ne peut prétendre à la justice, à la justesse et à l'égalité parfaites. Le système voulu par le Gouvernement laisse de côté tous ceux qui militent actuellement pour connaître leurs origines.

de la révélation de son identité à une personne issue de son don. Une telle idée méconnaît

que le donneur va avoir devant lui pendant toutes les années où l'enfant issu du don va grandir. Je recommande vraiment à nos collègues de s'en tenir à la formule de la commission

voire identifiantes. Je le rappelle, c'est une commission qui évalue les besoins de l'enfant et qui recontacte les donneurs. Il n'y a pas de mise en contact direct.

Je pense que c'est utile pour chacun. Ne troublez pas la qualité de ces débats en refusant de les donner. Ce serait dommage, madame la présidente.

Cela implique nécessairement une réflexion sur les procédures et les modalités concrètes de mise en oeuvre de cette faculté, qui, nous le savons tous, ne sont pas neutres. Le Gouvernement avait fait le choix, dans le texte initial, de recourir à la création d'une commission, pour assurer les missions d'accueil et de prise en charge des personnes nées d'une AMP avec don, ainsi que des tiers donneurs. Ce choix nous paraît plus pertinent que celui fait par la commission spéciale d'étendre les missions du CNAOP, aujourd'hui compétent pour l'accès aux origines des personnes nées sous X. Certes, le CNAOP est riche d'une expérience de plus de quinze ans en matière d'accès aux origines. Cependant, comme cela a été

Les débats de notre assemblée l'ont également rappelé : le recours à l'AMP avec tiers donneurs, d'une part, et l'adoption, d'autre part, induisent des réalités et des questionnements différents. Les enfants nés d'un don de gamètes et les enfants nés sous le secret n'ont pas un parcours et une histoire personnelle comparables. Réciproquement, l'implication d'un donneur ne peut être mise sur le même plan que celle de parents biologiques

différent de celui retenu par la commission spéciale, que je vous propose de rétablir à travers cet amendement. Il s'agit de confier à une commission, et non au CNAOP, les missions d'accueil et de prise en charge des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec don. a choisi de confier cette mission au CNAOP, qui intervient, je me permets de le rappeler, dans le cadre de l'accouchement dans le secret. Dans une première approche, le CNAOP pouvait sembler légitime pour remplir ce rôle, dans la mesure où son objectif essentiel est, en effet, de faciliter l'accès

selon nous un parallélisme infondé entre la situation des enfants nés dans le secret et celle des enfants nés d'une AMP avec tiers donneur. De même, le « don » de gamètes, conçu comme un acte solidaire et responsable, ne place en aucun cas le donneur dans une situation de dilemme ou de détresse assimilable à celle qui caractérise l'abandon d'enfant dans la situation particulière de l'accouchement sous le secret. Des effets délétères pourraient en résulter, tant pour les donneurs, en conférant une portée au don qui n'est pas légitime et qui peut constituer un frein à leur démarche, que pour les enfants nés d'une AMP avec tiers donneur, en suggérant que leur situation serait identique à celle des enfants relevant du CNAOP, avec finalement le risque de générer, par

Il est évident que ces deux régimes différents ne peuvent coexister, l'un permettant à des enfants d'avoir accès à leurs origines, l'autre ne leur permettant pas.

Au-delà des moyens supplémentaires à accorder aux Cécos, nous pensons qu'une des clés pour rendre réellement effective la PMA pour toutes est d'éviter la pénurie de gamètes. Quel est spéciale ? Vous avez bien compris que nous allons passer d'un système d'anonymat à un système qui lèvera, dans les conditions qui prévaudront à l'issue des discussions de ce texte, l'anonymat du donneur. Plusieurs phases sont prévues.

sur l'article. Le droit à l'AMP pour les couples de femmes ne saurait être pleinement effectif sans une reconnaissance juridique du lien de filiation entre l'enfant et ses deux mères et de la qualité de parents de ces dernières. Dans la suite logique de l'article 1, de loi consacre cette reconnaissance. Le mécanisme de la reconnaissance conjointe anticipée constitue, selon nous, la meilleure option parmi celles débattues en commission spéciale et, plus globalement, parmi celles avancées et discutées jusqu'ici dans le débat parlementaire.

de l'AMP, mais d'ajouter au régime de droit commun applicable aux couples hétérosexuels un régime spécifique pour les couples de femmes, ce qui ne permet pas, à notre sens, d'atteindre l'égalité. Des discriminations subsistent. Il serait dommage de ne pas les supprimer au moment, que l'on pourrait qualifier d'historique, où nous mettons fin à une grande injustice, en concrétisant le droit pour toutes à l'AMP. La première discrimination, c'est l'existence de deux modes d'établissement de la filiation distincts, selon qu'il s'agit d'un couple hétérosexuel ou d'un couple lesbien ayant eu recours à l'AMP. La deuxième discrimination, c'est l'absence de reconnaissance d'un lien de filiation, même en l'absence d'un lien biologique, par le mécanisme de la possession d'état pour les femmes concubines ou en couple ayant un enfant. La troisième discrimination, c'est l'absence de présomption de parentalité pour les couples lesbiens mariés, mécanisme reconnu pour les couples hétérosexuels mariés. Outre ces discriminations, nous regrettons que le mécanisme de reconnaissance de filiation conjointe anticipée soit entre les mains du notaire, et non entre celles du juge. Il s'agit d'un pas de plus vers la déjudiciarisation de tous les actes importants qui touchent au droit de la famille, processus que nous avons déjà dénoncé. Le groupe CRCE présentera des amendements visant à améliorer les dispositions de cet article afin, d'une part, de permettre la reconnaissance pleine et entière du lien de filiation entre l'enfant et ses deux mères sans qu'aucune discrimination subsiste dans la loi entre entre couples hétérosexuels et couples lesbiens et, d'autre part, de préserver les droits et l'intérêt de l'enfant, dont le mode de conception ne doit constituer ni une discrimination ni un obstacle à l'accès à ses origines. La parole

C'est la raison pour laquelle, en droit français et depuis toujours, la mère est la femme qui accouche. Il est très important que, au moment où nous voulons reconnaître une égalité de droits et de devoirs de deux femmes vis-à-vis d'un enfant qu'elles ont décidé de faire naître, nous n'abandonnions pas cette règle essentielle que je répète : la mère est la femme qui accouche. Par l'accouchement, on détermine un certain nombre d'obligations de cette femme vis-à-vis de l'enfant, puis, plus tard, de cet enfant vis-à-vis de cette femme. De mon point de vue, il n'est pas acceptable que l'on soit mère lorsque l'on accouche

l'égalité de droits entre les deux femmes en prévoyant que l'épouse ou la compagne de la mère sera autant mère que celle-ci, parce qu'elle aura bénéficié de la possibilité- ce sera même une obligation -d'adopter cet enfant selon une procédure automatique qu'elle ne pourra pas refuser. La parole est à M. Jacques Bigot,

n° 30 rectifié. L'article 4 tire les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et crée un nouveau mode de filiation fondé sur la volonté et détaché de toute référence à l'engendrement de l'enfant. Avec cette nouvelle rédaction, la filiation se détache du modèle biologique et n'a plus aucun rapport avec la réalité, puisque l'enfant pourrait, prétendument, avoir deux mères. Le principe selon lequel la femme qui accouche est la mère disparaît

qui n'est pas nécessaire. Il permettrait en effet d'établir la filiation, hors adoption, sur un pur critère de volonté de la part des deux mères, ce qui ne correspond pas aux principes fondamentaux du système français de filiation. Dans notre système, la filiation est établie selon le modèle de la procréation charnelle, qui implique qu'on puisse vérifier la réalité d'un lien de filiation, et il n'est pas possible d'utiliser ce modèle pour la femme qui n'a pas participé à la procréation charnelle.

Nous connaissons déjà l'adoption, qui, dans notre droit, est l'unique possibilité d'établir une filiation élective, c'est-à-dire une filiation sur la base de la seule volonté. Telle est la voie que nous proposons avec cet amendement ; il est un peu complexe et long, mais il est en réalité assez simple. Pour la femme qui accouche, nous ne changeons rien au droit existant ; ce serait toujours le seul accouchement qui entraînerait la maternité. Pour l'autre femme, celle qui ne participe pas à la procréation charnelle, l'amendement tend à instaurer une procédure d'adoption accélérée, dont le fonctionnement serait très simple. L'adoption serait ouverte à tous les couples, qu'ils soient mariés, concubins ou pacsés, comme le proposent d'ailleurs notre collègue Corinne Imbert et la députée Monique Limon. Le consentement à l'AMP chez le notaire vaudrait consentement à l'adoption,

le droit de la filiation. La commission spéciale n'a d'ailleurs pas procédé aux auditions nécessaires pour le faire. Nous ne sommes pas là non plus pour modifier la situation des couples qui ont aujourd'hui recours à l'assistance médicale à la procréation,

apporte quelque chose en matière tant de sécurité que d'égalité par rapport au schéma que l'Assemblée nationale a proposé. Voilà la raison pour laquelle il ne me semble pas opportun de recourir à la procédure judiciaire de l'adoption, comme vous l'imaginez. Je ne considère pas que votre proposition soit dénuée de sens,

ou contrainte supplémentaire aux femmes qui s'engagent dans ce processus. En quatrième lieu- nous l'avons rappelé à plusieurs reprises -, nous avons fait le choix de ne pas modifier

qui s'impose dans des conditions précisément fixées par la loi, selon des modalités très encadrées et avec des effets, eux aussi, précisément déterminés par la loi. Nous sommes vraiment dans un mode d'établissement de la filiation qui prend en compte la spécificité de cette situation, mais qui ne vient pas bouleverser le droit de la filiation. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne souhaite pas émettre un avis favorable sur l'amendement que vous portez, madame Primas.

pour dire que, dans la vie affective, dans la vie réelle de la famille à venir, deux femmes peuvent parfaitement élever un enfant,

On les cherche toute sa vie ! N'imposons pas aux enfants ces questionnements sur la façon dont ils sont venus sur Terre. Ils sont venus, parce qu'ils ont eu une maman. Cela ne remet pas en cause la place de la deuxième femme, qui peut l'aimer, l'adorer, mais cessons de vouloir trouver des solutions à un problème l'on ne mesure pas, que l'on ne maîtrise pas. Un enfant a toujours besoin de savoir. On ne ment pas à un enfant. On doit lui dire la vérité, même si elle est compliquée. Les adultes qui ont fait le choix d'être à deux mamans

chez les couples homosexuels que chez les couples hétérosexuels. Elle serait même plus forte chez les couples homosexuels féminins d'après les premières statistiques, mais nous n'avons pas encore suffisamment de recul. Pour ma part, je voterai l'amendement de Mme Primas,

cet acte fort que propose Mme Primas met les deux éléments du couple sur un pied d'égalité.

La PMA est possible. Pour autant, permet-elle à une femme qui n'a pas accouché de devenir mère ?

et ne pas mentir avec la réalité dans ces affaires extrêmement sensibles. Cela étant, l'amendement de Sophie Primas me paraît trop

La femme qui accouche est mère en toutes hypothèses, évidemment, mais elle serait mère célibataire, si je puis dire, s'il n'y avait cette reconnaissance conjointe qui bloque tout autre mode d'établissement de la filiation qui fera que les deux femmes seront mères en même temps. C'est un système extrêmement simple, clair, qui place les deux femmes à égalité. Il est respectueux du projet parental et me semble parfaitement s'inscrire dans la démarche que nous souhaitons promouvoir. Monsieur

le crois pas. À partir du moment où la filiation est établie, elle emporte exactement les mêmes conséquences, qu'il s'agisse de l'adoption, du système que nous proposons ou de la filiation biologique.

Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l'égard de chacune d'elles par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire. » Dans votre système, c'est donc la reconnaissance qui établit la filiation. Exactement ! Dissocier

: le Gouvernement ne conteste pas que, du point de vue de l'effet sur les droits et obligations des parents, l'amendement proposé par Mme Primas et la solution du Gouvernement ont exactement la même portée, à savoir que les deux femmes seront pleinement investies des droits et obligations d'une mère. C'est déjà très important, car tel est bien le principal objectif

doit être le même pour une femme qui accouche d'un enfant conçu avec un homme et pour une femme qui accouchera

aient exactement le même traitement juridique du point de vue de l'établissement de la filiation, dont j'ai essayé de rappeler tout à l'heure à quel point il était important qu'il repose sur des bases objectivement constatées, ! Par conséquent, tout le discours sur l'égalité et la discrimination se retourne complètement en faveur de la solution proposée par Mme Primas. L'adoption

la prudence. Si, chaque fois qu'un problème se pose, on remet en cause des modes d'établissement de la filiation maternelle établis depuis plusieurs siècles, on n'en sortira pas : ce sera la confusion dans l'établissement de la filiation maternelle

amendement ! J'espère, monsieur le président Bas, que vous reconnaîtrez que la solution proposée par le Gouvernement est préférable à la vôtre

Le scrutin est ouvert.

de la loi civile sur des situations déjà constituées poserait un problème de constitutionnalité. C'est une question très sensible en matière d'état des personnes.

mécanisme permet aux couples d'établir l'existence d'un lien de filiation avec leur enfant même en l'absence de lien biologique. Or, à ce jour, les couples de femmes ayant un enfant ne peuvent en bénéficier. Cela constitue une discrimination qui ne trouve aucune justification. Lors des auditions de la commission spéciale, nous avons pu entendre, notamment, les explications du porte-parole de l'Association des familles homoparentales, qui revendique l'ouverture de l'établissement de la filiation par la possession d'état

opposé. La mère sociale n'aura alors aucun moyen juridique de faire établir une filiation, même si elle a participé au projet parental et à l'éducation de l'enfant. Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette situation injuste et assez dramatique alors même que le projet de loi reconnaît aux couples de femmes le droit de construire un projet parental au même titre que les couples hétérosexuels. Nous proposons donc, par cet amendement de bon sens, de remédier à une injustice pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de ce texte et

à des couples de femmes sans établir de mode de filiation adéquat. Cependant, nous ne revisitons pas l'ensemble de notre droit de la filiation. Par ailleurs, outre les arguments que Mme la rapporteure a invoqués,

la possession d'état. Cette faculté lui serait ouverte pendant une période de dix années suivant la date à laquelle cette possession d'état aurait cessé en raison, notamment, de la séparation ou du décès.

nous dénonçons le caractère dérogatoire du régime de la filiation applicable actuellement aux couples lesbiens. En effet, nous ne voyons pas quel argument viendrait s'opposer à ce que les couples lesbiens mariés puissent prétendre au mécanisme de présomption de parentalité, sauf à créer une nouvelle fois une situation discriminatoire. Il s'agit ici d'une mesure de simplification et d'égalité. Quel est l'avis de la

La présomption de paternité est fondée sur le fait que, le couple étant marié et s'étant juré fidélité, dans les termes prescrits par le code civil, il est vraisemblable

Je vais donc suspendre la séance. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale à la prospective a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.